La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 6 novembre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ?

est, certes, une priorité, force est de constater les dérives de certains acteurs et les conséquences réelles de ce développement pour les riverains. Outre les démarches intrusives, les passages en force malgré les avis négatifs des communes, les utilisations sans autorisation de chemins communaux ou ou encore l'accaparement de parcelles communales, la multiplication anarchique des éoliennes mite inexorablement les paysages de cette région et exaspère la population. Or, à ce jour, la région Hauts-de-France remplit déjà ses objectifs pour 2020.

sur tout le territoire, et l'instauration d'enquêtes publiques internet, alors même que nos territoires ont de graves difficultés d'accès au réseau internet et que nombre de nos concitoyens sont frappés d'illectronisme, suscitent de grandes et fortes inquiétudes. Enfin, le

2 % de la production française ». En outre, dans les campagnes, le gigantisme des centrales éoliennes commence à détruire le corps social, entre ceux qui touchent de l'argent- propriétaires et collectivités -et ceux qui subissent les nuisances. Il paraît donc urgent de faire un état général des lieux des avantages et inconvénients des nouveaux modes de production d'énergie, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque ou la méthanisation, et d'associer effectivement et davantage les collectivités locales, les élus et les habitants aux projets ayant une incidence évidente sur leur quotidien. La parole

électrique français à moyen terme. Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, rendu public au début de 2019, confirme cette ambition. Vous l'avez indiqué, les objectifs fixés pour 2028 portent sur 15 000 mâts, soit moins d'un doublement par rapport à 2018. Les nouvelles installations sont plus efficaces et permettent de produire la même énergie que les anciennes avec un nombre plus réduit de mâts ; elles sont également moins coûteuses que par le passé. Le développement des projets éoliens est par ailleurs encadré par l'État. L'autorisation des projets relève du préfet et, dans ce cadre, on réalise une étude d'impact permettant la prise en considération de l'ensemble des enjeux. Une enquête publique est ainsi menée ; à ce titre, il est inexact de dire que le décret de décembre 2018 remplace l'enquête publique par une enquête électronique. Ce décret prévoit qu'une concertation en amont, sous l'égide d'un garant de la Commission nationale du débat public, doit être organisée, en respectant les conditions de transparence et de diversité des points de vue ; ce n'est qu'à cette condition que l'enquête électronique peut remplacer l'enquête publique traditionnelle. Toutefois, vous faites le juste constat que le développement de l'éolien, en France, est aujourd'hui porté en grande partie par la région Hauts-de-France. Cette réalité s'explique d'abord par les conditions favorables à ce développement : foncier disponible et ressources en vent. Ces différences géographiques, applicables à d'autres filières- photovoltaïque ou hydroélectrique, par exemple -, impliquent une participation à la transition énergétique nécessairement différente d'un territoire à l'autre, selon les ressources disponibles localement. Le Gouvernement est décidé à accompagner la filière éolienne, à l'améliorer, à oeuvrer dans le sens d'un développement accepté et maîtrisé de ce secteur, et ce avec l'appui précieux des régions. La parole est à M. Antoine

le secrétaire d'État, sur la nécessité de soutenir la réalisation d'un réseau express métropolitain dans le département d'Indre-et-Loire. Le projet de loi d'orientation des mobilités confirme la priorité donnée à la désaturation des villes et de leurs accès, ainsi qu'à l'amélioration des liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains. Ainsi, l'un des cinq programmes d'investissement porte sur la « résorption de la saturation des grands noeuds ferroviaires », avec pour objectif le doublement de la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. Pour ce qui concerne le traitement des noeuds urbains saturés, le rapport annexé au projet de loi prévoit d'engager 2,6 milliards d'euros dans les dix années à venir, hors Île-de-France, en associant l'État, les collectivités ou encore la SNCF. L'État y contribuerait à hauteur de 1,3 milliard d'euros. D'ici au 1 janvier 2020, SNCF Réseau doit soumettre à l'approbation du Gouvernement un plan d'ensemble précisant les objectifs visés, les les zones du réseau concernées par ce plan ainsi que les délais et les principales étapes de réalisation. Eu égard à sa position centrale et à la densité de ses lignes- dix branches ferroviaires, dont deux en ligne à grande vitesse -, le noeud ferroviaire de Tours-Saint-Pierre-des-Corps apparaît comme un point stratégique à l'échelon national. Il constitue également une réelle opportunité de promouvoir les mobilités décarbonées du quotidien. En effet, les onze intercommunalités du département sont innervées par les branches de l'étoile ferroviaire tourangelle et elles n'offrent pas moins de trente-trois points d'arrêt. Il existe donc une véritable possibilité de faire du ferroviaire une solution sérieuse de remplacement de l'automobile et un lien entre les territoires. Le 11 septembre dernier, le président de Tours Métropole et les présidents des dix communautés de communes du département vous ont sollicité afin que le bassin de vie tourangeau puisse devenir un terrain d'expérimentation du réseau express métropolitain. Aussi, je souhaite savoir dans quelle mesure le bassin tourangeau pourra être intégré à ce plan d'ensemble et, en particulier, si le Gouvernement entend soutenir le projet de réalisation d'un réseau express métropolitain dans le département d'Indre-et-Loire. La parole

appeler mon attention sur la réalisation d'un réseau express métropolitain dans le département d'Indre-et-Loire, notamment pour le noeud ferroviaire de Tours-Saint-Pierre-des-Corps. Vous l'avez rappelé, la priorité du projet de loi d'orientation des mobilités porte sur l'amélioration des transports du quotidien. En matière ferroviaire, il s'agit de doter les métropoles de liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées, à l'image du réseau express régional en Île-de-France, et d'élaborer, pour cela, un véritable schéma directeur pour des services express métropolitains. L'objectif est ambitieux : doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés,

mais le mode ferroviaire est encore largement sous-utilisé dans cette aire urbaine. SNCF Réseau a donc identifié l'étoile de Tours comme une zone de services potentiels de type « services express métropolitains », pour répondre à ces enjeux. Le plan d'ensemble, que doit présenter SNCF Réseau au début de 2020, permettra d'identifier les enjeux locaux et les leviers d'amélioration permettant de tendre vers la mise en place d'un tel réseau.

j'ai bien compris que, parmi les vingt noeuds métropolitains, le noeud de Tours et de la Touraine pourrait être bien placé. Les infrastructures existent, elles sont

Pendant plus d'un siècle, cette usine a fourni l'industrie française en zinc et en plomb. Elle a fait vivre des centaines de familles dans le Pas-de-Calais jusqu'à sa fermeture en 2003, mais elle a aussi pollué

Depuis lors, des centaines d'habitants ne peuvent plus disposer comme ils le souhaitent de leur propriété, certaines cultures sont impossibles et chaque projet d'urbanisme nécessite un décapage des sols très onéreux. Les élus de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et ceux des communes concernées ont donc décidé de réagir, en entamant une action demandant à l'État la réparation du préjudice écologique que subissent encore les populations et les collectivités du territoire En effet, l'État s'est contenté de constater les dégâts causés par l'ampleur de la pollution, mais il n'a pas pris toutes les dispositions pour l'éviter. Les élus locaux demandent donc aujourd'hui la prise en charge par l'État de la dépollution de l'ensemble des sols pollués. Cette mobilisation des élus de ce territoire, visant à mettre l'État face à ses responsabilités, me paraît d'autant plus légitime que ceux-ci ont l'impression d'être abandonnés par l'État. J'en veux pour preuve la non-compensation des exonérations de taxes foncières pour les propriétaires situés dans la zone du PIG, zone du PIG, compensation pourtant décidée par le Parlement en 2016. Le gouvernement actuel a décidé de ne pas honorer la parole de l'État, ce qui occasionne, pour les collectivités concernées, une perte financière d'un million d'euros et engendre des difficultés budgétaires importantes pour nombre d'entre elles. Je souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement au sujet de cette situation insupportable, à l'origine des actions légitimes des élus locaux qui se battent pour le respect de leur territoire. La parole Monsieur le ministre, qui concerne la pollution causée par l'ancienne usine Metaleurop Nord, sachez que le ministère de la transition écologique et solidaire est, depuis de nombreuses années, actif sur ce dossier complexe et sensible. En effet, avant même la fermeture de l'usine, des dispositions ont été prises, au titre de la réglementation des installations classées, conduisant à réduire fortement les émissions dans l'air et dans l'eau. Ainsi, grâce à l'action des services de l'État, les rejets atmosphériques en plomb ont été divisés par au travers notamment d'un contrat signé en 2003 avec la région, les conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, et les présidents des trois communautés d'agglomération, à la reconversion industrielle du site, pour aider au reclassement des anciens salariés. Cette reconversion, d'un budget de 66 millions d'euros, a fait l'objet d'un accompagnement public de 14,1 millions d'euros. Afin de prévenir les risques sanitaires et environnementaux liés à la pollution des sols, des restrictions d'urbanisme ont été instaurées

l'enlèvement des terres et matériaux pollués chez les particuliers, un accompagnement à la reconversion des parcelles agricoles touchées et la protection des cours d'école. Ces mesures ont été mises en oeuvre dès la fermeture de l'usine. Par ailleurs, M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, avait apporté, lors de la séance du 20 novembre 2018, une réponse à votre question relative à la non-compensation des exonérations de taxes foncières, qui relève de son ministère.

Ces terres de travail, qui souffrent encore de l'après-mine et de la pollution à tout crin, déplorent aujourd'hui l'abandon de l'État, qui n'assume pas ses responsabilités. Je prends acte de vos éléments de réponse, mais je ne me résigne pas à les accepter pour solde de tout compte. La

dans bien des domaines, lequel territoire en aurait grandement besoin. Face à ce pillage incessant, et qui n'est pas sur le point de se terminer, il existe une production légale qui, au contraire, diminue d'année en année, et qui représente désormais à peine par an. Cela est dû à des tracasseries administratives, trop souvent infondées, à une obstruction administrative quasi systématique, qui, étant très souvent proche de l'arbitraire, Est-ce la manifestation d'une politique masquée visant à arrêter l'exploitation légale ? C'est la question qui se pose avec encore plus d'acuité depuis qu'ont été portés à notre connaissance les premiers éléments de la réforme du code minier. Ces éléments sont très inquiétants et mettent en émoi, en ébullition, toute la profession légale, qui existe depuis longtemps et qui doit maintenant se battre pour exister. Cela, vous semblez l'ignorer ou n'en faire que peu de cas. L'inquiétude est donc très vive dans la profession, car la future procédure d'instruction des demandes de titres miniers prévue dans votre projet de réforme sera plus complexe, alors que, déjà, les délais actuels de traitement se situent entre quatre et Pourquoi ne pas intégrer un délai légal de réponse de l'administration, au-delà duquel un accord tacite serait accordé, comme cela se fait dans d'autres domaines ? Enfin, que dire de la possibilité de refuser un titre minier pour un motif environnemental, motif non défini avec précision dans votre projet de réforme ? s'agit-il pas là d'une porte ouverte à un refus systématique de toute demande et d'un moyen non avoué de tuer le secteur minier ? Monsieur le secrétaire d'État, j'attends une réponse claire, ferme et définitive du Gouvernement à ma question

La réforme du code minier que le Gouvernement promeut s'inscrit dans la continuité des travaux et des concertations antérieurs, et dans une volonté que les projets miniers autorisés soient à la hauteur de nos ambitions en matière environnementale. Plus particulièrement, ce projet entend prendre en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des territoires dès les premières autorisations. L'objectif est d'aboutir à des procédures plus transparentes, à des décisions plus protectrices de l'environnement et à des modalités de participation du public renforcées, tout particulièrement pour les titres de recherche, et ce préalablement aux premières demandes de travaux. Par ailleurs, cette révision des procédures d'autorisation ne sera pas nécessairement plus longue, si l'ensemble des parties prenantes sont consultées bien en amont des décisions.

une fédération, la Fédération départementale d'énergies des Ardennes ; ce syndicat intercommunal à vocation multiple est l'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie dans le département. À ce titre, cette fédération, qui regroupe l'ensemble des communes ardennaises, assure le maintien et le développement d'un réseau électrique de qualité dans le département, mais participe également au déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques et à la réalisation de la cartographie numérique du territoire.

du développement des énergies renouvelables au sein des communes, ainsi que pour les opérations visant à faciliter la transition énergétique. Dans ces conditions,

Les syndicats d'énergie jouent un rôle déterminant dans la qualité de la distribution d'énergie, au travers de leurs investissements dans les réseaux, mais ils sont également des acteurs majeurs de la transition énergétique locale, en accompagnant le développement des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et de la maîtrise de l'énergie.

En particulier, des dispositions ont été prévues par le Gouvernement pour permettre aux syndicats de prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Le Gouvernement a également souhaité étendre le champ d'intervention du financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale, outil de péréquation indispensable dont bénéficient de nombreux syndicats. La parole est à M. Marc Laménie,

Mme Loisier appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la représentation des entreprises du secteur éolien au sein de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (Ofate). Cet organisme est supposé coordonner les politiques franco-allemandes. À cet effet, il a ses bureaux dans les locaux mêmes du ministère, et il est financé, pour plus d'un tiers, par celui-ci. Son comité de pilotage est notamment composé des quatre syndicats d'énergies renouvelables franco-allemands, et nombre des autres membres ont des intérêts particuliers de ce secteur. Il semble donc que le lobby éolien soit financé par le ministère lui-même ... Par ailleurs, le rapport franco-allemand d'Agora Energiewende et de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) indique que, « si des capacités nucléaires sont retirées du mix français, la compétitivité des centrales à charbon maintenues dans le système en Allemagne est améliorée ». L'Allemagne aurait donc doublement intérêt à ce que la France renforce ses capacités de production d'énergie éolienne, car non seulement elle compte de nombreuses entreprises dans ce secteur, mais en outre la baisse des capacités nucléaires françaises rendrait plus compétitifs les centrales à charbon et leur maintien en Allemagne. Mme Loisier demande donc à Mme la ministre son analyse sur ces faits au regard des intérêts de la France en matière de politique énergétique. La parole

dans le but de promouvoir l'information et la coopération entre les deux pays concernant l'ensemble des énergies renouvelables. L'Ofate n'a pas de mission de coordination des politiques énergétiques de la France et de l'Allemagne. Il s'agit d'une association visant à partager et à échanger. Par ailleurs, l'éolien ne constitue qu'une partie du travail de l'Ofate, qui couvre également le photovoltaïque, les bioénergies, les questions de marché et de réseaux électriques, l'efficacité énergétique et la chaleur. Pour répondre à ses missions, l'Ofate a été créé dans un format mixte public-privé, et il est financé partiellement par les ministères français et allemand chargés de l'énergie et par ses membres issus du monde de l'énergie. Les publications de l'Ofate sont publiques et visent à éclairer toutes les parties prenantes, ainsi que le grand public, sur les conditions juridiques, techniques et économiques de la transition énergétique dans les deux pays et de mettre en relation ces parties prenantes à tous les échelons. La coopération franco-allemande dans le domaine énergétique, permise en partie par l'Ofate, constitue un atout pour la transition énergétique en ce qu'elle permet une meilleure diffusion des connaissances, des retours d'expériences internationaux et des évolutions. Enfin, l'Ofate n'a pas participé à l'élaboration du rapport Agora-Iddri que vous avez mentionné. La conclusion que vous citez est l'un des résultats de cette étude, qui se projette dans un marché européen surcapacitaire, dans lequel la France et l'Allemagne auraient développé les énergies renouvelables tout en maintenant leur parc de production conventionnelle. Or un tel scénario ne paraît plus d'actualité compte tenu notamment des annonces allemandes relatives à la sortie du charbon dans la production d'électricité, avec la fermeture de centrales pour un total d'environ 12 gigawatts d'ici à 2023.

sa perplexité quant au choix de la France de réduire ses capacités nucléaires au point, peut-être, de menacer sa sécurité d'approvisionnement. Au reste, ce choix donne raison au maintien, par l'Allemagne, de ses centrales à charbon, ce qui, sur le plan environnemental, est particulièrement déconcertant.

Monsieur le secrétaire d'État, le 27 mai dernier, en votre qualité de corapporteur de la mission d'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, vous avez effectué, en train, le trajet Grenoble-Veynes. Au mois de septembre dernier, dans les colonnes du, vous avez tenu des propos qui se voulaient « rassurants », confirmant la volonté de l'État de sauver l'étoile de Veynes, en prenant en charge une partie des travaux. Pourtant, malgré les déclarations de bonnes intentions et les financements annoncés, notamment par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, métropole grenobloise et les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère et de la Drôme, bien qu'ils n'en aient pas la compétence, les élus nationaux, locaux et les usagers ne sont pas entendus. En effet, en décembre 2020, SNCF Réseau suspendra l'exploitation de la ligne des Alpes n° 905, faute d'investissements. C'est à la même période que seront effectués les travaux de modernisation et de sécurisation des voies sur la section Livron-Veynes. Cela revient à dire, monsieur le secrétaire d'État, que le département des Hautes-Alpes, malgré ses 140 000 habitants, ses 387 000 lits touristiques et ses 20 millions de nuitées par an, n'aura tout simplement plus de desserte ferroviaire, ni par Grenoble ni par Valence. Je souhaite donc connaître très clairement la position de l'État sur ce dossier et surtout savoir si vous avez l'intention ou non de prendre la main pour que SNCF Réseau lance enfin

Celle-ci participe, en effet, à la vitalité des territoires des Alpes du Sud, tout en les reliant aux Alpes du Nord, facilitant ainsi les échanges entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je partage entièrement votre préoccupation quant à sa pérennité. Sur la section entre Grenoble et Vif, des travaux sont prévus en 2020 pour éviter une fermeture. En revanche, les circulations sur la section Vif-Veynes devraient être suspendues en décembre 2020, faute d'entretien lourd depuis des années.

à décembre 2021, la branche Livron-Veynes sera fermée pour travaux, afin d'assurer, pour l'avenir, la pérennité de l'axe ferroviaire reliant Valence à Briançon et, ainsi, le maintien des circulations du train de nuit Paris-Briançon. Une offre de substitution au train de nuit sera également mise en place en 2021, pendant les travaux. Le Gouvernement a demandé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réunir un nouveau comité de pilotage d'ici à la mi-décembre 2019, afin d'étudier avec les collectivités locales les propositions actualisées de SNCF Réseau et d'organiser un tour de table sur les questions financières. En tout état de cause, madame la sénatrice, soyez assurée que l'État veillera à ce que les solutions permettant de pérenniser la desserte des Hautes-Alpes soient mises en oeuvre dans les meilleures conditions pour les usagers du train.

visant l'obtention du baccalauréat parallèlement à la pratique intensive d'une discipline sportive à haut niveau. C'est le cas, par exemple, de nombreux skieurs, comme ceux du lycée de Villard-de-Lans dans mon département, mais cela concerne aussi d'autres parcours de formation destinés à des sportifs de très haut niveau. Ces élèves ont une scolarité aménagée, qui leur permet de mener à bien leur double projet sportif et scolaire. La promotion inscrite depuis 2018, qui n'est donc pas concernée par la dernière réforme du baccalauréat, passera cet examen en juin 2021, soit l'année du premier nouveau baccalauréat réformé. Depuis un an, ces élèves sont bien préparés au baccalauréat actuel, et certains ont même d'ores et déjà passé des épreuves. Aujourd'hui, la décision concernant les conditions d'obtention finale de leur baccalauréat n'est toujours pas définie. Le double projet est pourtant une politique sportive et éducative ambitieuse, largement soutenue par le Gouvernement. Aussi, il paraît nécessaire de sécuriser le parcours de ces jeunes sportifs, en leur permettant de passer des épreuves alignées avec les programmes actuels. Cette solution apparaît aujourd'hui comme la plus raisonnable pour nos sportifs de demain et répond avant tout à une question d'égalité. Une proposition a été soumise au rectorat de Grenoble, initiative fondée sur le travail en commun des inspecteurs, proviseurs et enseignants. Cette proposition est, à ce jour, restée sans réponse. ministre, quelle est votre position à ce sujet ? Que comptez-vous faire pour permettre à ces jeunes de ne pas être pénalisés dans leurs parcours scolaire et sportif ? Il est urgent de rassurer ces adolescents et leurs familles, alors même que la saison d'hiver va débuter et que d'importantes épreuves vont

pleinement emparée de la situation particulière des 143 élèves skieurs sportifs de haut niveau bénéficiant d'un étalement du cycle terminal sur trois années scolaires. Du fait des aménagements de scolarité prévus pour leur permettre de concilier scolarité et entraînement sportif, ces élèves ont suivi les deux premiers trimestres de l'année de première

élèves passeront leurs épreuves finales du baccalauréat lors de la session 2021. Ils relèvent donc du baccalauréat général et technologique tel qu'il vient d'être réformé. Ce cas est prévu par la réglementation du nouveau baccalauréat. Les élèves skieurs de haut niveau de l'académie de Grenoble pourront ainsi, comme tous les sportifs de haut niveau, bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, lequel permet aux élèves sportifs de haut niveau de valider leur contrôle continu par le biais d'épreuves ponctuelles, à la fin de l'année de terminale, sur autorisation du recteur d'académie. Ils auront bien fait, comme tous les autres candidats scolarisés de la session 2021 du baccalauréat, une année de terminale « rénovée », ce qui leur permettra de présenter les épreuves terminales, celles de spécialité, comme celle de philosophie, ainsi que le grand oral. Il est vrai que, au titre du contrôle continu, ces élèves sont supposés se présenter à une épreuve commune pour l'enseignement de spécialité qu'ils n'ont pas poursuivi en classe de terminale. Après étude de la situation présentée par Mme la rectrice, il apparaît que l'organisation de la scolarité de ces élèves ne leur permet pas de préparer cette épreuve commune de contrôle continu pour l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale dans les meilleures conditions. Afin de répondre à cette situation, un arrêté sera publié prochainement, prévoyant, pour tous les élèves bénéficiant d'un aménagement de scolarité permettant que leur année de première se déroule sur les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, une dispense de l'épreuve commune de contrôle continu pour l'enseignement de spécialité suivi en première, mais non poursuivi en classe de terminale. Cette dispense concerne uniquement l'épreuve ; elle n'est donc pas une dispense d'enseignement. À ce titre, l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale sera pris en compte dans la note de bulletin pour l'année de première. Ces aménagements témoignent du bon niveau d'adaptation de la réforme du lycée et du baccalauréat aux différentes situations rencontrées par les élèves : même si celles-ci concernent un petit nombre d'élèves et des cas très particuliers, nous pouvons parfaitement adapter la scolarité. Monsieur le

environ 400 000 se trouvent en situation de handicap : enfants avec trouble du spectre autistique, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, adolescents dyspraxiques ou dyslexiques ... Tout élève reconnu handicapé et ayant besoin d'un accompagnateur doit avoir à ses côtés un AESH pour lui permettre de mener sa scolarité le mieux possible. Chaque rentrée scolaire apporte toutefois son lot de problèmes : enfants sans accompagnants, accompagnants sans affectation, établissements scolaires non prévenus de l'arrivée d'un AESH La dernière rentrée ne fait pas exception puisque, depuis le mois de septembre dernier, plus de 200 AESH, dans la seule académie de Rouen, travaillent sans contrat de travail ou sans salaire, voire les deux à la fois. Certains accompagnants n'ont, à ce jour, toujours pas reçu leur affectation. Cette situation plonge les accompagnants d'élèves handicapés dans une grande précarité. Le travail qu'ils réalisent auprès des enfants et adolescents en situation de handicap est pourtant essentiel. Il est incompréhensible que ces professionnels, dont le rôle est d'assurer l'inclusion de toutes et tous au sein de l'école de la République, travaillent bénévolement ou soient empêchés de remplir leur mission, alors que les enfants et adolescents en situation de handicap ont besoin d'eux. Notre système est capable d'assurer, chaque année, la rentrée scolaire de 12 millions d'élèves. Il est inacceptable qu'il ne sache assurer celle des 400 000 élèves en situation de handicap et qu'il contrevienne ainsi au principe selon lequel le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction. à l'heure où l'inclusion de personnes en situation de handicap a été érigée comme l'une des priorités du quinquennat du Président de la République, comment expliquez-vous ces graves dysfonctionnements ? Sont-ils liés à la mise en place, à la rentrée, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, dont l'un des objectifs était pourtant de professionnaliser les accompagnants et d'améliorer leurs conditions de travail ? Quelles mesures votre ministère entend-il prendre pour remédier à ces problèmes et éviter qu'ils ne se reproduisent à la rentrée prochaine ?

enregistrés dans l'académie de Rouen. La rentrée a vu la création d'un service de gestion dédié aux accompagnants dans les directions départementales des services de l'éducation nationale et dans les rectorats, de façon justement à déprécariser les personnels en charge de l'accompagnement des élèves handicapés.

de déprécarisation. Compte tenu des règles de la comptabilité publique, les agents qui ont été recrutés au début du mois de septembre n'ont pas tous pu bénéficier d'une rémunération complète au titre du mois de septembre dès la fin dudit mois : la paie de septembre étant clôturée,

Pour les dossiers qui n'étaient pas complets aux échéances de transmission, il n'a pas été possible de s'appuyer sur cette procédure. Il s'en est ensuivi que certains AESH n'ont pas pu percevoir de rémunération, ce qui est évidemment tout à fait anormal. Saisi de ces situations, le ministère s'est rapproché des services de la direction générale des finances publiques pour permettre que soient transmises au comptable, dès lors que les dossiers de prise en charge étaient complets, des demandes d'acompte en dehors des dates fixées par le calendrier national. Ainsi, pour l'académie de Rouen, le versement d'acomptes s'est poursuivi sur les mois d'octobre et de novembre. Un pilotage renforcé permettra de parvenir à une régularisation de ces situations dans les meilleurs délais. Bien entendu, chacun sera désormais payé en temps et en heure.

de trois ans a permis des progrès, mais il faut aller vers une professionnalisation encore plus grande de ces agents de la fonction publique et leur offrir, à terme, des contrats à durée indéterminée.

Ce Camsp accueille plus de 260 enfants en situation de handicap, dans le but que ceux-ci puissent vivre sereinement et s'intégrer dans la société. Pour ces enfants et leurs familles, il est un acteur absolument indispensable. Pourtant, depuis 1993, le personnel du Camsp du Mans exerce dans des locaux préfabriqués inadaptés. Cette situation, censée être provisoire, perdure depuis plus de vingt ans. Les locaux, devenus de surcroît insalubres, ne sont plus aux normes. Pour exemple, les entrées ne sont même pas accessibles aux fauteuils roulants : un comble pour un établissement d'accueil de personnes en situation de handicap ! Par ailleurs, le nombre de demandes de prise en charge par le Camsp ne cesse d'augmenter chaque année. Malgré ces difficultés, les professionnels du Camsp demeurent très investis et motivés, en trouvant des expédients plus ou moins efficaces. Ainsi, les personnels n'hésitent pas à partager leur bureau à chaque nouvelle intervention pour pouvoir recevoir un enfant supplémentaire. De même, en mai 2018, le personnel du Camsp du Mans avait monté un projet d'achat de nouveaux locaux, avec un plan d'investissement, à l'attention de (ARS). Voilà un an et demi que le personnel du Camsp attend une réponse, alors que la situation presse. La ministre des solidarités et de la santé ainsi que la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées ont toutes deux insisté sur l'importance de la prévention et ont réitéré cette priorité dans le cadre du plan Autisme 2018-2022, afin de favoriser le diagnostic précoce. Au regard de la motivation et du dévouement réel des équipes que j'ai rencontrées, il est urgent

L'amélioration tant de la qualité de l'accueil des familles que des conditions de travail des professionnels constitue une priorité et un engagement constant des services de l'ARS comme de ceux du conseil départemental de la Sarthe,

L'ARS Pays de la Loire a réuni, le 2 octobre dernier, les acteurs concernés, à savoir, l'association gestionnaire du Camsp, le conseil départemental de la Sarthe et le centre hospitalier du Mans, afin de discuter à nouveau des enjeux et de la situation. Une méthode de travail a été retenue. Le principe de la relocalisation du Camsp sur le site de l'hôpital du Mans et d'un soutien au Camsp qui implique la réalisation de travaux de restructuration des bâtiments du centre hospitalier du Mans, permet d'envisager, selon le calendrier prévisionnel, une implantation dans de nouveaux locaux en septembre 2021. Il appartient désormais à l'association gestionnaire de formaliser l'expression de ses besoins de la maîtrise d'ouvrage, en vue de finaliser le projet architectural et de définir le schéma de financement associé. Enfin, pour répondre aux besoins immédiats du Camsp, à savoir

Or les conditions de travail relèvent plus que jamais de l'enjeu plus global de santé publique, parce qu'elles concernent la préservation de la santé de ces personnels, dans un environnement de travail particulièrement pathogène, à fort taux de pénibilité et dont les contraintes sur les organismes sont lourdes de conséquences. Or, vous le savez, madame la secrétaire d'État, le secteur hospitalier pâtit d'un manque notoire de personnels. L'hôpital n'attire plus non plus les étudiants. Enfin, des études démontrent clairement que le manque durable de personnels engendre des désorganisations importantes au sein de la majorité des hôpitaux français. Les personnels hospitaliers, dans leur grande majorité, sont confrontés à de telles contraintes que leurs effets délétères sur la santé ont été montrés du doigt par les épidémiologistes. Comment maintenir la qualité des soins dans cet environnement de travail de plus en plus difficile et dans ce contexte de manque d'effectifs véritablement problématique ? Madame la secrétaire d'État, depuis des mois, les établissements publics de santé sont secoués, partout, par des mouvements sociaux sans précédent, notamment au sein des services d'urgences, de maternité, de la protection de l'enfance, des structures pour personnes âgées et dans les secteurs de la psychiatrie. Tous dénoncent le manque de moyens matériels, humains, budgétaires et la souffrance au travail. Quelle part

de nos soignants. L'amélioration des conditions de travail des hospitaliers est une condition nécessaire pour maintenir la qualité des soins et préserver l'attractivité de nos hôpitaux. C'est aussi et avant tout quelque chose que nous devons aux hospitaliers qui, chaque jour, soignent nos concitoyens. Vous l'avez rappelé, des tensions sociales s'expriment dans des établissements de santé depuis plusieurs mois. Les problématiques qu'elles recouvrent ne datent pas d'hier, mais il est de notre responsabilité d'y répondre. Tout d'abord, une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail a été lancée pour faire de ce sujet une priorité. Plusieurs des mesures de cette stratégie sont déjà en place. L'Observatoire national de la qualité de vie au travail a été installé. Il a pour mission de recueillir et de capitaliser sur les données existantes de manière à améliorer le suivi de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Il nous fera des recommandations pour que de nouvelles actions soient déployées. Ensuite, un dispositif de médiation à l'échelle nationale et interrégionale est en cours de déploiement : les médiateurs seront susceptibles d'intervenir à la demande des établissements ou des professionnels pour mener des conciliations, notamment dans le cadre de conflits en lien avec les conditions de travail. Par ailleurs, depuis deux ans, le Gouvernement a pris des mesures importantes pour apporter des solutions concrètes à ces difficultés. Pour la première fois en dix ans, les tarifs hospitaliers ont été augmentés en 2018 et de nouveaux moyens pérennes ont été alloués à la psychiatrie. Nous avons mis en oeuvre une stratégie de transformation du système de santé, intitulée qui comprend des mesures importantes pour soutenir les établissements de santé et accompagner les carrières des professionnels de santé, qu'ils soient en exercice ou en formation. Plusieurs mesures illustrent notre ambition à agir pour mieux accompagner les professionnels et rendre les métiers plus attractifs. Les études médicales sont, par exemple, en train d'être réformées pour arrêter le gâchis humain de la sélection en fin de première année et la compétition excessive des épreuves classantes nationales avant l'internat. Des travaux sont également en cours pour adapter les parcours professionnels des hospitaliers, notamment afin de leur permettre de diversifier

Je vous remercie, Il y a urgence à agir, en particulier sur les territoires ruraux, confrontés au problème de l'accès aux services sanitaires. Les hôpitaux sont souvent, à cet égard, le premier et dernier recours dans ces territoires. La parole

et de la santé. Madame la ministre, depuis septembre 2018, l'assurance maladie rembourse les téléconsultations faites un ordinateur, un smartphone ou une tablette, mais elle limite le remboursement à celles qui sont réalisées auprès du médecin traitant ou d'un médecin ayant une connaissance préalable du patient. Si les téléconsultations se développent, leur progression est beaucoup plus lente que prévu. Le Gouvernement en prévoyait 500 000 pour 2019 et 1 million en 2020, mais ce sont à peine 60 000 qui ont été constatées après un an, alors qu'il y a 350 millions de consultations physiques. Ce démarrage timide s'explique par de nombreuses barrières. La pratique, en outre, concerne majoritairement l'Île-de-France. Seulement 1 600 médecins libéraux ont facturé des actes en télémédecine cette année et certaines plateformes n'arrivent même pas à obtenir le remboursement des actes par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), sous divers motifs. Pourtant, la téléconsultation permet de désengorger les services médicaux d'urgence. Elle permet aux patients d'avoir accès à un médecin, qu'il soit leur médecin leur médecin traitant ou non. Il n'y a pas de raison de pénaliser les malades qui font l'effort de ne pas se déplacer aux urgences, en ne les remboursant pas ! En outre, compte tenu de la nécessité pour les médecins et les utilisateurs de disposer d'une connexion internet suffisamment bonne

que représente son déploiement. Les pratiques médicales et soignantes à distance constituent une opportunité majeure dans l'organisation de notre système de santé et pour l'amélioration de l'accès aux soins. Pour ces raisons, le Gouvernement a permis une accélération sans précédent de son déploiement, avec l'entrée dans le droit commun de la tarification des actes de téléconsultation et de téléexpertise, et la création du télésoin dans le cadre de « Ma santé 2022 Vous interrogez le nombre d'actes de télémédecine depuis la mise en place du remboursement. Le nombre de 60 000 actes de téléconsultation est un indicateur, mais l'étude de la progression du nombre d'actes mensuels est davantage révélatrice du dynamisme de la télémédecine

Leur répartition doit donc s'observer au regard de la démographie régionale. Vous mentionnez des barrières à la télémédecine. Celles-ci peuvent être surmontées. Il s'agit d'une évolution culturelle très importante. À ce titre, beaucoup a déjà été fait. À la demande d'Agnès Buzyn, la Haute Autorité de santé a édité un guide de bonnes pratiques en télémédecine, notamment en téléconsultation. Des formations sont mises en place dans le cadre du développement professionnel continu et des discussions sont en cours pour l'intégration dans la formation initiale. Par ailleurs, l'encouragement aux usages se poursuit avec la création, pour les infirmiers, d'un acte d'accompagnement du patient à la téléconsultation. Il est également prévu de prendre en charge l'accompagnement à la téléconsultation des patients par le pharmacien en officine. L'application de ces mesures sera effective dès janvier 2020. Vous mentionnez enfin la nécessité d'une couverture numérique satisfaisante pour la mise en oeuvre de ces nouvelles pratiques. Les objectifs du Gouvernement sur ce sujet sont donc un bon débit pour tous et la généralisation d'une couverture mobile de qualité dès 2020 et du très haut débit pour tous en 2022. Comme vous le voyez, de nombreuses mesures sont déjà mises en oeuvre. Nous continuerons de mettre en place des actions permettant le déploiement d'organisations de télémédecine et l'accès des patients à cette innovation. La parole

ont déjà consommé de l'alcool, 44 % d'entre eux ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois et près de 9 % ont une consommation régulière d'alcool. Ces chiffres appellent à reconsidérer en profondeur les politiques de prévention, en particulier celles qui visent à protéger la jeunesse. Mais notre socle législatif en la matière semble bien en peine. Les alcooliers débordent d'imagination pour contourner la loi Évin : « marques alibis » pour parrainer des événements destinés aux jeunes, publicité directe- toujours pour viser les jeunes -des influenceurs sur les réseaux sociaux ... Les exemples illustrant la nécessité de compléter cette loi ne manquent pas. Face à un constat que nous partageons sans doute, vous avez préféré confier la prévention aux alcooliers eux-mêmes. Nous avons alors vu apparaître les campagnes d'apprentissage au goût conduites par les alcooliers auprès de très jeunes enfants et d'adolescents. Sous couvert d'une volonté de jouer un rôle préventif, les alcooliers font valoir qu'une « bonne éducation » dans l'enfance protège de tous les excès de consommation à l'âge adulte. D'importants moyens de communication sont déployés au moyen de kits pédagogiques, de jeux s'adressant à des enfants de 4 à 14 ans, visant à leur faire découvrir l'univers de la vigne, les goûts et les terroirs. Cet « apprentissage du goût » dès le plus jeune âge favoriserait un comportement responsable chez les adultes « avertis » de demain

se réfèrent à la tradition. La science, elle, appuyée par de nombreuses études, montre que cette prétendue « éducation à bien boire » est en réalité une incitation à boire. Comment Comment comptez-vous mettre enfin un terme à ces pratiques en contradiction totale avec les objectifs de santé publique ? Qu'envisagez-vous pour créer un réel environnement protecteur pour notre jeunesse où l'alcool ne serait pas ainsi banalisé ? La parole

mais surtout qu'elle favorise les comportements ultérieurs à risque, à la fin de l'adolescence. Une chose est sûre avec la molécule d'alcool, c'est son caractère toxique sur les cellules cérébrales des enfants et adolescents.

La découverte du patrimoine et la promotion de l'alcool sont deux choses différentes. Jean-Michel Blanquer, qui est aussi engagé pour la santé des jeunes, a eu l'occasion de rappeler aux recteurs d'académie que toutes les précautions nécessaires devaient être prises en cas d'utilisation de ces kits du fait des risques d'incitation à la consommation d'alcool et de banalisation de son usage qu'ils pourraient présenter. Des messages de prévention et d'information sur les risques doivent y être systématiquement associés. La promotion des comportements favorables à la santé auprès des jeunes est essentielle. Nous avons notamment lancé le service sanitaire des 48 000 étudiants en santé et inscrit l'« école promotrice de santé » dans le

je me vois contrainte de vous la poser à nouveau, en présence, d'ailleurs, des salariés de l'établissement. La situation s'aggrave. L'ensemble des services est touché. Il ne s'agit plus seulement du service de soins de longue durée. Le manque de médecins est une des causes de ces dysfonctionnements et fermetures de lits. Or aucune annonce n'a été faite. Le dispositif de recrutement choisi par la direction- « activer le réseau » -est un échec : 9 médecins ont démissionné en raison de la dégradation des conditions de travail.

et n'est donc plus reconnue en tant que telle. La pérennité de l'unité de soins palliatifs est remise en question depuis le départ d'un médecin en juin 2019 et d'un autre en fin d'année. Le service d'addictologie a vu la fermeture de 6 lits sur 22 par manque de médecins. L'hôpital de jour du service nutrition-obésité fonctionne au ralenti avec un demi-service fermé depuis depuis août dernier. Depuis le mois de septembre, il ne reste qu'un médecin pour les quatre services de long séjour de 179 lits. La direction a décidé d'en réduire le nombre à 90 lits. lits. Lorsque tous les lits sont ouverts, ils sont occupés. Dorénavant, les patients sont mis à la porte de l'hôpital. Au regard de la démographie des personnes âgées, l'heure serait plutôt à l'augmentation de lits en gériatrie plutôt qu'à leur fermeture ... Que dire alors du projet du Gouvernement d'admettre directement les personnes âgées en service de médecine gériatrique pour leur éviter les urgences ? Pour couronner le tout, madame la secrétaire d'État,

Il y a eu des départs de médecins dans la plupart des disciplines représentées sur le site- gériatrie, soins palliatifs, addictologie. Le groupement hospitalier a mis en oeuvre les procédures de recrutement, mais le contexte actuel de pénurie dans certaines spécialités médicales, comme la gériatrie, induit un délai de recrutement incompressible. En dépit de ces difficultés, la communauté médicale de René-Muret s'est mobilisée pour restreindre autant que possible les fermetures. L'institution s'appuie sur une stratégie interne de recrutement et de publication afin de maintenir une offre de soins dans un département fragile. hôpital joue un rôle essentiel dans les soins prodigués en proximité aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Ses activités médicales ne sont nullement remises en question. Au contraire, le projet stratégique de l'hôpital en cours de discussion vise à renforcer le service rendu aux usagers. Ces difficultés de recrutement sont prises en compte avec une stratégie de transformation de l'offre, en particulier sur les soins de longue durée. La prise en charge sanitaire devrait évoluer en faveur d'une augmentation de lits de SSR neurologiques, d'une création d'un hôpital de jour et de lits supplémentaires de SSR polyvalents. S'agissant des soins de longue durée à l'hôpital René-Muret, le site offre aujourd'hui des conditions d'hébergement vétustes, en inadéquation avec les besoins des personnes âgées, qu'il est indispensable de faire évoluer. Pour autant, il y a non pas une réduction des capacités de prise en charge, mais une transformation de l'offre pour consolider la filière gériatrique. Des échanges ont eu lieu cet été sur l'évolution du site avec les représentants syndicaux de l'hôpital, les représentants de l'AP-HP et de la délégation départementale de l'ARS Sur le sujet majeur de l'attractivité du site pour les professionnels de santé, les évolutions prévues sont de nature à en améliorer le positionnement dans la filière de soin du territoire et à améliorer les conditions de travail dans un cadre architectural rénové. Enfin, sur les métiers de la gériatrie, l'AP-HP travaille à offrir des perspectives d'évolution et de carrière aux professionnels en prévoyant notamment, dès 2020, le déploiement de la formation d'assistant de soins en gérontologie auprès de 300 aides-soignants. La parole

participer à un essai clinique. Ces soins peuvent être pris en charge par la sécurité sociale, mais ils représentent des coûts très importants pour des chances de réussite moindres, l'état des enfants s'étant encore aggravé en raison du temps perdu pour faire les démarches et de la fatigue du voyage.

Au mois de janvier dernier, nous avons demandé, avec une centaine de mes collègues sénateurs, que les cancers de l'enfant et de l'adolescent soient déclarés grande cause nationale pour 2019. Il y avait certainement des sujets plus importants puisque nous n'avons pas été entendus

secrétaire d'État. Madame la sénatrice, ce sujet dont vous souhaitez qu'il obtienne le label de grande cause nationale tient particulièrement à coeur à la ministre Agnès Buzyn, qui a eu l'occasion de le rappeler ici à plusieurs reprises. Nous partageons évidemment votre souhait de renforcer notre politique de lutte contre les cancers pédiatriques. Il appartiendra au Premier ministre de se prononcer le moment venu sur cette labellisation. Soyez assurée que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question. La lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent est en effet une priorité. C'est le sens des actions portées par le plan Cancer III. Elle constituera sans nul doute un des axes importants de la future stratégie décennale de lutte contre le cancer, prévue par la loi du 8 mars dernier relative aux cancers pédiatriques. L'effort de recherche français sur les cancers pédiatriques, réalisé dans le cadre des deux premiers plans Cancer, représentait 10 % du financement de la recherche publique en cancérologie. Sous l'égide des ministères en charge de la recherche et de la santé, l'Institut national du cancer (INCa) y consacre à ce jour plus du tiers de ses recettes, soit environ 100 millions d'euros. Une attention particulière a été accordée aux avancées de la recherche fondamentale en cancérologie avec l'affectation de moyens publics augmentés, en 2018, de 5 millions d'euros Par ailleurs, la loi du 8 mars 2019 permet de nombreuses avancées, notamment en matière de soutien aux aidants familiaux par le recours à un nouveau congé de présence parentale et de prise en charge de la douleur, en particulier par les centres d'oncologie pédiatrique, par l'évaluation de l'efficacité des moyens dédiés et par le renforcement de la formation des professionnels de santé dans ce champ. Une avancée majeure en faveur des patients concerne le droit à l'oubli. Un rapport du Gouvernement au Parlement est prévu sur l'application de la convention Aeras- -pour préciser les possibilités d'évolution du dispositif pour une prise en compte des pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de 21 ans et un accroissement des sanctions en cas de manquements à la convention. à la convention. Nos efforts pour réduire les effets de la maladie sont de plus en plus efficaces. L'amélioration de l'accès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes aux solutions médicales les plus innovantes demeure un enjeu majeur

secrétaire d'État, vingt-cinq hôpitaux d'Île-de-France ont failli fermer leurs urgences pédiatriques, faute d'internes en nombre suffisant. Cette situation vient du fait que la répartition des internes de médecine générale dans les différents services de pédiatrie de la région

santé (ARS), les résultats de la procédure de choix des internes de médecine générale pour le semestre d'hiver 2019 ont conduit non seulement à une réduction du nombre d'internes ayant choisi d'effectuer leur stage dans un service de pédiatrie, mais surtout à une répartition de ces 159 internes qui n'est pas en adéquation avec les besoins de fonctionnement des services de pédiatrie et d'urgences pédiatriques : 327 postes ont postes ont été ouverts, mais seulement 159 internes les ont choisis, dont une écrasante majorité pour des postes à Paris et en petite couronne, délaissant ainsi les établissements de grande couronne. ces derniers se sont retrouvés sous-dotés en interne, alors que le semestre d'hiver est le plus chargé en raison des épidémies de bronchiolites, de grippes, de gastro-entérites, etc. Au final, le directeur de l'offre de soins de l'ARS a trouvé une parade en relançant la procédure de choix de ces internes à la faveur d'un incident constitutif d'une atteinte au principe d'égalité. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous affirmer que le risque de fermeture des urgences pédiatriques est définitivement écarté ? Alors que ces services sont déjà pénalisés par le manque de pédiatres en raison d'une démographie défavorable et du manque d'attractivité des carrières hospitalières,

l'issue de la première procédure de choix des internes de médecine générale laissait craindre de fortes tensions dans de nombreux services de pédiatrie de petite et de grande couronne du fait d'une répartition des internes qui n'était pas en adéquation avec les besoins de fonctionnement de ces services. Plusieurs pistes ont fait l'objet de discussions avec l'ensemble des parties prenantes. La mise en évidence d'un problème de conformité lors de la première procédure de choix a conduit l'ARS Île-de-France à relancer en urgence la procédure. la procédure. La commission de répartition s'est de nouveau réunie le 22 octobre dernier pour proposer un nombre de postes ajusté, une répartition plus équilibrée et plus pertinente, ainsi que des mesures de soutien aux internes affectés par ce changement. Les nouveaux choix ont été faits le mardi 29 octobre, en accord avec les internes et leurs représentants : 182 internes ont choisi le stage de médecine générale en pédiatrie pour le semestre d'hiver 2019, contre 159 lors de la première procédure,

comme chaque semestre, des postes restent vacants dans certains établissements, le nombre de postes ouverts étant réglementairement supérieur au nombre d'internes susceptibles de les choisir. Sur les territoires en situation de fragilité, notamment dans le nord des Yvelines, les organisations territoriales devront être adaptées, avec le soutien de l'ARS. Enfin, conformément aux engagements pris par l'ARS, les par l'ARS, les 267 internes ayant changé de lieu de stage entre le premier et le second choix bénéficieront d'une prime exceptionnelle de 400 euros par mois durant toute la durée de leur stage. La parole est

stricte de l'obligation de débarquement : exemption, exemption pour haut taux de survie autorisant le rejet de certaines espèces dans des pêcheries identifiées, flexibilité interzonale, flexibilité interespèce ... Ce travail s'est fait avec les représentants des

des anciens rejets de poissons ayant la taille commerciale et désormais inclus dans le calcul des TAC. Nous faisons tout pour essayer de répondre positivement aux contraintes et aux demandes des pêcheurs.

entre pêcheurs amateurs installés sur les bords des gaves d'Oloron et de Pau et pêcheurs professionnels qui exercent leur activité dans l'estuaire de l'Adour. Deux points de vue s'opposent dans un climat de moins en moins serein. pêche, supposée trop forte, empêcherait le saumon de remonter les gaves. Les associations de pêcheurs amateurs et de défense de l'environnement dénoncent un risque pour le renouvellement de l'espèce et les maires de la communauté de communes Béarn des Gaves une menace sur une filière touristique majeure. Gestion rigoureuse, pratiques vertueuses et déclaration systématique de la totalité des captures, les pêcheurs professionnels répliquent que la menace sur le renouvellement de l'espèce relève du fantasme et que les règles sont respectées. Le 25 juin dernier, en l'absence d'une autorisation du concessionnaire du port, à savoir le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le tribunal administratif de Pau enjoignait le préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en oeuvre son pouvoir de police pour que la pêche aux filets dérivants dans le port de Bayonne cesse. En aucun cas, la décision de la juridiction administrative ne se fondait sur une analyse de la gestion des stocks. En juillet, le comité interdépartemental des pêches publiait une étude selon laquelle le stock de saumons en migration dans l'Adour se portait bien et ne nécessitait pas de mesures de gestion supplémentaires. Monsieur le ministre, pour vous qui étiez venu au port de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure voilà un an jour pour jour et qui connaissez bien ce territoire et ses acteurs, il n'est pas besoin de grands mots pour comprendre la difficulté de la situation. Déjà, en avril, je vous demandais qu'une étude indépendante soit mandatée par l'État afin d'objectiver la situation en termes de ressources, d'atténuer ces tensions croissantes et de rétablir un peu de sérénité. Au regard des derniers événements, je renouvelle ma demande. Pouvez-vous vous engager à ce qu'une étude objective soit lancée afin de déterminer dans quelle mesure le renouvellement du saumon est réellement menacé dans l'Adour et dans les gaves ? La parole

juin dernier, une décision de justice a interdit la pêche dans le port de commerce de Bayonne. Le tribunal exige des préfets qu'ils fassent appliquer les dispositions du code de transport interdisant la pêche dans les ports de commerce, sauf

commission administrative compétente pour régler les usages et organiser la concertation. Ces acteurs locaux mettent en oeuvre la gestion des pêcheries de saumon, dans le cadre des directives internationales de l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord et de la réglementation nationale. Si je le précise, c'est parce qu'il y a des contraintes et des règles incontournables. incontournables. Vous soulevez le besoin d'information pour apaiser les tensions entre les pêcheurs amateurs et les pêcheurs professionnels, et vous avez entièrement raison. Je pense qu'il faut renforcer nos connaissances scientifiques pour objectiver la situation de l'état des stocks.

En 2018, des milliers de mètres cubes de bois ont dû être abattus dès les premiers signes d'attaque et mis en vente. Mais l'afflux massif de résineux a fait baisser des deux tiers le prix moyen du mètre cube. Malheureusement, l'hiver 2018-2019 a été clément, et l'été 2019 encore plus chaud et sec que celui de 2018. Aujourd'hui, l'Office national des forêts (ONF) parle de centaines de milliers de mètres cubes de bois à traiter, soit des dizaines de milliers d'arbres à couper au plus vite et à commercialiser. C'est une véritable tempête silencieuse. Le volume est d'ailleurs supérieur à celui qui avait été constaté à l'issue des tempêtes de Noël 1999. Cependant, il n'y a aucun moyen de lutter efficacement contre cet insecte, vivant sous l'écorce des arbres, si ce n'est un hiver froid et des arbres capables de se défendre en produisant de la sève et des terpènes à haute concentration, s'ils ne souffrent pas de stress hydrique. Vous en conviendrez, à l'avenir, ces conditions d'absence de sécheresse et de froid hivernal risquent d'être plus difficiles à réunir. Aussi, dans plusieurs articles de presse, l'ONF annonce à court ou moyen terme la disparition de tous les résineux dans les forêts situées à moins de 500 mètres d'altitude. En outre, la disparition des résineux entraîne une fragilisation de l'ensemble du biotope forestier. Ainsi, de nombreux feuillus souffrent à leur tour de l'assèchement du sol consécutif à la disparition des résineux et, stressés, sont eux aussi sensibles à différentes attaques. Les frênes de Moselle sont touchés par la chalarose, les hêtres, particulièrement sensibles à la sécheresse, souffrent beaucoup et meurent également nombreux. En Moselle, le président des communes forestières,

Aujourd'hui, du producteur au transformateur scieur, toute la filière bois est profondément touchée. L'État n'est pas en reste, puisque nous sommes propriétaires collectivement de près de 70 % des forêts du Grand Est, et donc touchés par cette catastrophe. Aussi, monsieur le ministre je voudrais savoir quelles mesures d'urgence vous comptez mettre en place pour accompagner la filière, notamment les propriétaires publics comme privés, face à ce désastre sanitaire, au-delà des 16 millions d'euros débloqués dernièrement et bien insuffisants selon tous les acteurs.

du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Les directives nationales visent à une scolarisation en milieu ordinaire d'au moins 80 % des mineurs avec troubles du comportement. Il s'agit de sortir les mineurs des établissements relevant de l'agence régionale de santé pour un hébergement avec une scolarisation en établissement classique. L'ARS a souhaité que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) signent une convention pour mettre en oeuvre le dispositif d'interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques (ITEP). Celui-ci permet aux directeurs des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques de sortir les mineurs de leur structure pour qu'ils restent à domicile avec intervention d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). La MDPH du Jura a refusé de signer cette convention. En effet, la mise en oeuvre d'une telle disposition aura des conséquences financières majeures pour les conseils départementaux. Ces directives vont dans le bon sens, puisqu'elles facilitent l'intégration des enfants handicapés, et les collectivités s'organiseront en conséquence. Toutefois, les conseils départementaux s'inquiètent de l'augmentation des dépenses obligatoires liées à l'application de ces mesures.

la réponse qu'elle m'a transmise. Il n'y a pas de report de charges sur les collectivités dans le cadre du fonctionnement en dispositif ITEP (Ditep). Permettez-moi de redire que nous devons garantir aux personnes en situation de handicap une participation pleine et entière à l'exercice de leur citoyenneté. Pour répondre à cette exigence, si légitime, les politiques publiques du handicap ont pris une orientation résolument inclusive, dans la continuité des avancées portées par la loi du 11 février 2005, la grande loi sur le handicap voulue par le président Chirac. D'une manière générale, la mise en oeuvre d'une politique inclusive repose sur deux principes fondamentaux : d'une part, l'appui sur les ressources du milieu ordinaire, que ce soit l'école, le logement, l'emploi ou encore la santé ; d'autre part, l'appui sur l'évolution des pratiques d'accompagnement mises en oeuvre par les opérateurs médico-sociaux, dont l'expertise, importante et tout à fait nécessaire, doit permettre de rendre possible le choix des personnes, selon des solutions adaptées. Ce dernier point n'inclut nullement la disparition des moyens médico-sociaux existants. Il vise à les déployer de manière différenciée au plus près des besoins des personnes et selon une capacité d'intervention graduée. Le fonctionnement en Ditep s'inscrit complètement dans cette orientation. Ce dispositif favorise une meilleure prise en charge des besoins des jeunes vers le milieu ordinaire. Il s'adresse à un public présentant des difficultés psychologiques, mais dont les capacités cognitives sont préservées, et vise à faciliter les passages entre les modalités d'accompagnement proposées par les ITEP et les Sessad, sans devoir repasser par les MDPH-

En Bourgogne-Franche-Comté, une convention DITEP régionale a été signée en 2018 par l'ensemble des partenaires signataires obligatoires de la convention, à l'exception de la MDPH du Jura et de la MDPH de la Côte-d'Or, et ce malgré le travail partenarial mené depuis 2018 avec les MDPH, l'ARS, les services académiques, les organismes de protection sociale et les gestionnaires d'ITEP et Sessad. Un comité stratégique du parcours handicap assure le suivi de la mise en oeuvre de la convention et élargira le périmètre de celle-ci aux conseils départementaux, à la protection judiciaire de la jeunesse et à la pédopsychiatrie. Aussi, je ne peux qu'inviter la MDPH du Jura à rejoindre ce dispositif conventionnel, dont la réussite est très largement saluée. Telle est, madame la sénatrice, la

Le conseil départemental du Jura m'a fait part des nouvelles charges induites par cette mesure. La liste des charges transférées ou imposées aux conseils départementaux sans compensation suffisante est lourde. Sans contester le bien-fondé de la mesure de scolarisation des mineurs en situation de handicap en milieu ordinaire, il convient au minimum d'évaluer et de compenser les nouvelles charges induites pour les conseils départementaux. La parole

de fabrication de pneumatiques Bridgestone situé à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Depuis un an, l'attitude du groupe japonais laisse craindre le pire. A-t-il l'intention de fermer le site de Béthune, qui emploie encore plus de 1 000 salariés ? Dès le début des années 2000, le groupe a développé ses activités en Europe de l'Est, dans des usines largement financées par l'Union européenne. Il continue à y consacrer l'essentiel de ses investissements. Dans le même temps, il met en concurrence ses sites d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est celui de Béthune qui est malheureusement visé par cette logique. Accusé d'être le moins rentable du groupe, il est privé des investissements nécessaires à sa modernisation. Dans un contexte où le marché est en crise, comme en atteste l'annonce de la fermeture de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon, la direction de Bridgestone a décidé de ramener le « ticket », c'est-à-dire l'objectif de production, de 18 000 pneus par jour en en 2018 à 9 000 à la fin de l'année 2019. Une centaine d'emplois intérimaires est en passe d'être supprimée. Je sais que le Gouvernement n'est pas sans rien faire. Même le Président de la République a échangé sur ce sujet avec le Premier ministre japonais au printemps dernier. Plus récemment, plusieurs réunions à haut niveau se sont tenues, à Bercy, avec M. Paolo Ferrari, président européen du groupe. Mais rien ne transpire de ces échanges. Ce silence contribue à installer une psychose

été particulièrement suivi par le Gouvernement, qui avait salué l'accord collectif de performance trouvé fin avril-début mai, grâce d'ailleurs à l'action de ses services et aux nombreux contacts qui ont été pris, y compris avec l'actionnaire japonais. Aux termes de cet accord, l'actionnaire s'engageait à investir massivement sur le site et à préserver les quelque 1 000 emplois du site. Cet accord a été soumis à un référendum des salariés. Il a malheureusement été rejeté. Il est particulièrement regrettable que des informations parfois erronées aient été relayées au moment de la présentation de cet accord de performance collective, alors même qu'une issue positive aurait permis la réalisation d'investissements nécessaires sur le site, l'assurance d'une charge correcte de l'usine jusqu'en 2021 et une garantie de l'emploi associée. Un accord aurait été aussi utile pour démontrer à la direction japonaise la volonté de toutes les parties prenantes d'aller de l'avant. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons maintenu le contact avec l'actionnaire Bridgestone. J'ai moi-même saisi M. Ferrari, que vous avez évoqué. Sans cet accord, nous sommes dans une conjoncture délicate. Le marché du pneumatique en France et en Europe est particulièrement difficile

Les échanges se poursuivent entre la direction et mes équipes, en liaison avec la région Hauts-de-France. À ce stade, aucun des éléments transmis par les actionnaires ne permet d'affirmer que le groupe Bridgestone souhaite fermer l'usine de Béthune. En tout état de cause, nous sommes mobilisés aux côtés des salariés et des élus du territoire pour donner à l'entreprise un avenir. J'appelle donc chacun à prendre ses responsabilités pour que le site renoue avec un climat social apaisé permettant de trouver une issue avec l'actionnaire japonais. La parole

Madame la secrétaire d'État, depuis de trop nombreuses semaines, la distribution du courrier dans le Val-de-Marne est sujette à d'importantes difficultés. Ces problèmes, qui étaient déjà sensibles depuis quelques mois, se sont profondément aggravés ces derniers temps, avec, au mois de septembre, des quartiers entiers non distribués et de nombreux plis non acheminés. Quand les courriers arrivent enfin, ce n'est pas toujours chez le bon destinataire. Cette situation a pénalisé aussi bien les habitants que les entreprises. Comme prise de paralysie, La Poste n'a, encore à ce jour, adressé aucune information aux usagers. Le contrat d'entreprise entre l'État et La Poste pour 2018-2022 a été signé en janvier 2018. Celui-ci lie l'État à La Poste pour la bonne exécution des des quatre missions de service public confiées par la loi à celle-ci, dont le service universel postal courrier et colis fait partie. À cet effet, l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques définit les contours contours du service universel, qui comprend notamment une levée et une distribution six jours sur sept sur l'ensemble du territoire national. Le contrat entre l'État et La Poste n'a pas été respecté. Face aux carences dans la distribution du courrier postal, l'engagement, la mobilisation et la détermination des maires et de leurs équipes municipales sont entiers. Il y a un an déjà, nombre d'élus locaux, dont M. Olivier Capitanio, maire de Maisons-Alfort, Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont, ou encore Metin Yavuz, conseiller départemental à Valenton, étaient mobilisés devant le ministère de l'économie pour rappeler au Gouvernement le rôle crucial d'un service public postal. Mme Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, et M. Patrick Beaudouin, maire de Saint-Mandé, également échangé avec la direction de La Poste. Les municipalités ont ainsi mis en relation La Poste avec tous les acteurs locaux, afin de faciliter les résorptions de ses problématiques d'emploi. Aux côtés des élus locaux, nous avons convenu que l'opérateur transmettrait un état hebdomadaire de l'évolution de la situation, et notamment des moyens qu'il mettait en oeuvre pour résorber les courriers en souffrance, chiffres à l'appui. En fin de semaine dernière, La Poste indiquait que seulement 40 % des courriers en souffrance dans la commune de Vincennes étaient traités et qu'elle espérait un retour à la normale pour la fin du mois. C'est une évolution positive, mais nous restons mobilisés et particulièrement inquiets quant à la concrétisation des efforts engagés par La Poste.

prendre pour nous garantir que La Poste respecte scrupuleusement le contrat de service public universel qui la lie à l'État, dans le Val-de-Marne comme sur l'ensemble du territoire national ? La parole est à

le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'État est particulièrement attentif. La distribution du courrier relève du service universel postal. L'État veille à ce qu'elle soit réalisée dans le respect des objectifs de de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise et traduits dans des arrêtés annuels, ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public- vous l'avez précisé. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de distribution est du ressort de La Poste. Elle représente un enjeu majeur pour l'entreprise, qui doit notamment s'adapter à la réduction des volumes de courrier à traiter. Vous le savez, l'activité traditionnelle de La Poste, à savoir le transport et la distribution du courrier, se réduit de manière inexorable. Les volumes de courrier adressés sont en baisse drastique depuis plus de dix ans : ils sont passés de 17,7 milliards d'objets en 2008 à 9,9 milliards d'objets en 2018, soit- 43 % en dix ans, à raison d'une baisse de 7 % par an. La Poste réorganise son réseau de distribution, tout en développant de nouvelles activités, pour s'adapter à l'évolution des besoins des usagers des services postaux et répondre à leurs attentes en matière de services de proximité et de croissance du marché des colis et marchandises. Pour continuer à assurer ses missions de service public, tout en préservant son modèle social, La Poste a fait le choix stratégique d'investir sur l'atout majeur de son réseau de factrices et de facteurs. Toutefois, dans le Val-de-Marne, l'entreprise connaît des difficultés récurrentes de recrutement et de fidélisation des facteurs, notamment sur le bassin d'emploi où se situe le site de Vincennes. En effet, de grands chantiers se préparent en Île-de-France - le Grand Paris, les jeux Olympiques de 2024, la remise à niveau de certaines infrastructures, la construction de 70 000 logements -, qui captent une large part du marché de l'emploi. Pour faire face à cette pénurie de recrutement, La Poste s'efforce de trouver au plus vite des solutions en s'appuyant sur ses partenaires locaux. Les nouvelles organisations nécessaires à la transformation de La Poste se mettent en place, en tirant profit des progrès progrès réalisés en termes de mécanisation du tri et de préparation par tournée des sacoches de distribution des facteurs. Dans le Val-de-Marne, comme dans les autres départements, la mise en place de ces nouvelles organisations a nécessité un temps d'adaptation pour les agents. Ainsi, après de nécessaires ajustements, une nouvelle organisation de la distribution postale a pris effet le 16 septembre dernier au centre courrier en charge de Vincennes et de Saint-Mandé. Pour autant, en dépit des plans de formations et de l'accompagnement des personnels pour assurer la continuité du service public, ces nouvelles organisations ont généré dans les premiers temps des difficultés dans la distribution du courrier. Interrogée sur les carences signalées à Vincennes en particulier, La Poste affirme qu'elle est très attentive aux perturbations qui affectent la distribution du courrier et qu'elle déploie depuis plusieurs semaines un plan de retour à la normale. À l'échelle

simplifiée, et que ces Américains accidentels puissent pleinement bénéficier des possibilités de régularisation rapide de la situation fiscale qu'offre le droit américain. remboursement de la dette sociale (CRDS) avait été finalement réglée par un accord entre les deux administrations fiscales. Le fisc américain a par ailleurs décidé d'accorder un dégrèvement aux personnes ayant renoncé à leur citoyenneté américaine depuis le 18 mars 2010, sous certaines conditions. En revanche, il semble qu'aucune avancée n'ait été enregistrée s'agissant de la transmission du numéro d'identification fiscale (NIF) américain. Craignant des sanctions, les banques françaises ont fait savoir qu'elles pourraient être contraintes de mettre fin aux relations commerciales qu'elles entretiennent avec des « personnes américaines », autrement dit

Ce constat est particulièrement inquiétant ; il concerne 40 000 de nos concitoyens. Je souhaite donc savoir si les démarches entreprises par le gouvernement français auprès des autorités de Washington ont des chances d'aboutir d'ici au 31 décembre. La parole est à Mme la secrétaire

une décision juridique sur la position que nous défendions, selon laquelle la CSG et la CRDS constituent des impôts, couverts à ce titre par la convention fiscale qui lie nos deux États. Cette inflexion permet de résoudre des situations préjudiciables de double imposition. ailleurs, l'(IRS) a présenté le 6 septembre dernier une nouvelle procédure d'amnistie fiscale. Celle-ci constitue une avancée significative qui, compte tenu des seuils de référence élevés, permettra de résoudre la situation fiscale de nombreux binationaux ayant décidé de renoncer à leur nationalité américaine. S'agissant des problématiques rencontrées par les clients de nationalité américaine dans leurs relations avec les établissements bancaires, consécutives aux difficultés de délivrance, par les autorités américaines, d'un numéro de sécurité sociale qui fait également fonction de numéro d'identification fiscale- le (TIN) -,

Les représentants parlementaires ont été amenés à insister auprès des responsables du Trésor américain sur l'urgente nécessité de résoudre ces difficultés. Nous avons nous-mêmes beaucoup échangé avec l'administration américaine et ces initiatives viennent d'aboutir à la publication par l'IRS, le 15 octobre dernier, de compléments aux instructions existantes qui précisent les obligations des institutions financières en matière de collecte et de transmission du TIN. Or ces instructions amendées reconnaissent désormais expressément que, après l'échéance du 31 décembre 2019, le défaut de transmission d'un TIN par les banques n'emporte nullement pour conséquence immédiate la caractérisation d'un manquement significatif de leur part. Les services de l'IRS prendront en considération les circonstances particulières ayant conduit à cette carence, ainsi que les procédures internes mises en place et les diligences accomplies par les institutions financières pour collecter cette information. Théoriquement, à compter du 1 janvier 2020, les citoyens

commune. La procédure est laborieuse : le maire doit mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de réparer le véhicule et de recourir pour ce faire à un expert automobile qui doit déterminer si le véhicule est réparable ou non. Cette étape franchie, le maire peut procéder à la mise en fourrière du véhicule ou à son évacuation d'office vers un centre de véhicules hors d'usage agréé. Mais la question qui se pose trop régulièrement est : qui prend en charge le financement de l'ensemble de ces opérations conduites par le maire lorsque le propriétaire du véhicule est insolvable, injoignable ou inconnu ? Ces cas, malheureusement les plus fréquents, ne sont pas clarifiés par le droit en vigueur. En toute logique, le dernier propriétaire de la carte grise enregistrée sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) devrait être tenu de régler la facture à la place de la collectivité. Tel était le sens de l'amendement que j'avais présenté dans le cadre du projet de loi Engagement et proximité. Le Gouvernement l'a balayé d'un revers de main au motif que cet amendement était « satisfait ». Satisfait, pourtant, personne ne semble l'être ! L'accès au SIV est autorisé aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route or certaines dispositions relatives à la gestion des épaves de voitures relèvent du code de l'environnement. Il y a donc un problème de concordance et d'application des codes. En outre, si le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, bénéficie d'un accès direct à cette plateforme, il peut manquer de formation ou d'information ; or les agents de l'administration des finances publiques, eux, n'ont qu'un droit de transmission indirect restreint.

Ce flou législatif et réglementaire a un coût. Ce coût est par exemple, pour Bordeaux, de 226 euros par véhicule, après une procédure extrêmement chronophage. Cette procédure est également décourageante pour beaucoup de maires qui ne peuvent plus ou pas s'acquitter de cette charge financière.

lorsque le propriétaire du véhicule s'est avéré inconnu, introuvable ou insolvable. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas adapté de faire peser sur le dernier détenteur du certificat d'immatriculation du véhicule la charge de s'acquitter de l'avance des frais de fourrière, alors que celui-ci n'est plus le propriétaire dudit véhicule, qu'il a cédé a cédé légalement. Néanmoins, les frais de fourrière représentant un coût important pour les autorités dont relèvent les fourrières, la Délégation à la sécurité routière développe un système d'information national des fourrières automobiles pour limiter ce coût et moderniser et moderniser les procédures applicables. Ce système devrait être opérationnel à la fin de l'année 2020 et les collectivités territoriales pourront y adhérer. S'agissant de l'accès au système d'immatriculation des véhicules, que vous sollicitez, l'article L. 330-2 du code de la route l'ouvre déjà aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences, ainsi d'ailleurs qu'aux agents de police judiciaire adjoints, aux gardes champêtres et aux maires. Les modalités d'accès aux informations contenues dans le SIV sont suffisantes, en l'état, pour permettre le recouvrement forcé des frais engagés. Toutefois, ce sont les ventes frauduleuses de véhicules d'occasion ainsi que le non-respect des obligations liées à l'immatriculation des véhicules par certains propriétaires qui rendent parfois complexe,

Madame la secrétaire d'État, je veux attirer votre attention sur le statut des forestiers-sapeurs. Ces fonctionnaires territoriaux principalement chargés de la surveillance des massifs forestiers, de la réalisation des travaux d'entretien

ils contribuent au signalement des feux naissants et combattent les incendies au péril de leur vie. Sur le terrain, qu'ils connaissent parfaitement, ils ont un rôle essentiel et indispensable. Bien qu'ils aient obtenu des évolutions de leur statut, avec une reconnaissance de leurs compétences professionnelles, le métier de forestier-sapeur n'est pas référencé par le répertoire des métiers territoriaux élaboré par le Centre national de la fonction publique territoriale. La catégorie d'emploi retenue dans le cadre de la prise en compte de la pénibilité au travail et dans le calcul de leurs pensions de retraite est la catégorie sédentaire,

La prise en compte de la pénibilité de certains métiers devait faire l'objet d'une réflexion d'ensemble dans le cadre de la réforme des retraites. Mais cette réforme aura-t-elle lieu avant quarante ans ? Les forestiers-sapeurs seront alors tous grands-pères, mais à la retraite

Ce classement se traduit par l'établissement d'une liste réglementaire d'emplois, qui se compose des emplois publics afférents à certains grades et corps expressément énumérés. Le bénéfice de ce classement peut en outre être conditionné à la satisfaction de critères spécifiques, tels que le critère du « contact direct et permanent avec des malades » ou le fait d'occuper l'emploi auprès d'une administration donnée ou dans un domaine donné. Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, le classement dans la catégorie active n'est pas retenu. Pour les agents affiliés à la CNRACL, ce classement est actuellement établi par l'arrêté du 12 novembre 1969 modifié. Eu égard à l'organisation actuelle de la fonction publique territoriale par cadres d'emplois, les fonctions effectivement exercées au sein d'un même cadre d'emplois peuvent donner accès ou non, selon leur nature, aux avantages liés à la catégorie active, dont le bénéfice est apprécié par les services gestionnaires de la CNRACL. À cet égard, l'arrêté du 12 novembre 1969 précité prévoit le classement dans cette catégorie des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que de certains ouvriers professionnels dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles, et qui sont expressément listés dans l'arrêté. Ces emplois correspondent dorénavant à ceux auxquels peuvent être affectés les adjoints techniques territoriaux, par exemple. Bien que les emplois de forestiers-sapeurs puissent également être occupés par des adjoints techniques territoriaux, ils ne font pas expressément partie de la liste établie par l'arrêté précité. Le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier cet arrêté pour en étendre le champ de manière ponctuelle. En effet- vous l'avez dit -, la prise en compte des risques et de la pénibilité de tel ou tel emploi ne peut désormais être traitée indépendamment de la réflexion transversale et globale- et actuelle ! -qui est menée sur la pénibilité par le haut-commissaire aux retraites. Et, comme vous le savez, nous parlons là de décisions qui doivent aboutir en 2020, et certainement pas dans

En réponse aux questions écrites que nous avons adressées à M. le ministre, ses services sont restés pour le moins évasifs ; ils s'abritent derrière le secret fiscal, alors que les comptes de l'Agedi, établissement public gestionnaire de deniers publics, sont publics. Cela n'a aucun sens. Par ailleurs, les autres arguments invoqués par l'administration sont totalement infondés. Tout d'abord, le Gouvernement justifie l'assujettissement de l'Agedi à l'impôt sur les sociétés par le fait que le syndicat ne répondrait pas à un besoin fondamental des populations. Or la jurisprudence limite cette exigence aux cas où il existe une régie, ce qui n'est pas le cas pour l'Agedi. Il paraît tout de même aberrant, en outre, de prétendre que doter une mairie de moyens informatiques nécessaires à son bon fonctionnement, à l'heure de la dématérialisation des services, ne répondrait pas à un besoin collectif des populations. Enfin, si l'on reprend la fameuse règle des « 4 prix, produit, public, promotion -, vos services ne peuvent, comme ils le font, prétendre que l'activité de l'Agedi serait lucrative et indistincte de celle des éditeurs privés. Ses adhérents n'acquittent à aucun moment un prix qui incorporerait une marge, et l'Agedi ne fournit pas de matériel. Les collectivités membres de l'Agedi sont, dans leur immense majorité, des collectivités de petite taille qui ne disposent ni du budget nécessaire ni du personnel possédant les compétences informatiques requises et l'Agedi ne procède à aucune démarche de promotion commerciale. Il est ainsi clair que ce syndicat n'exerce en aucune façon son activité dans les mêmes conditions que les acteurs privés de l'édition de logiciels. Ce positionnement de l'administration fiscale ne dissimule-t-il pas, madame la secrétaire d'État, la volonté politique d'une nouvelle ponction fiscale sur des collectivités, souvent parmi les plus pauvres, leurs syndicats ?

en vertu du secret fiscal, nous ne communiquons pas d'informations relatives à la situation fiscale particulière d'un contribuable. Vous savez d'ailleurs que des discussions approfondies sur le traitement de l'Agedi sont en cours entre

résulte de la nature des activités qu'elles exercent. Ainsi, ces personnes morales, telles que les syndicats mixtes, sont soumises aux impôts commerciaux lorsqu'elles exercent une activité lucrative, c'est-à-dire une activité concurrentielle réalisée dans des conditions similaires à celles qui président pour le vérifier, comme vous l'avez dit, les produits proposés, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée. Même lorsque le critère de lucrativité est satisfait, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités peuvent, conformément à une jurisprudence constante, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés si les services rendus sont indispensables à la satisfaction des besoins collectifs de la population, notamment en raison d'une carence de l'initiative privée. La détermination du régime fiscal applicable suppose donc l'examen, cas par cas, de la nature des activités exercées et de leur mode d'exploitation. C'est ainsi que nous procédons. Par respect

Toutes les charges de fonctionnement d'un Ehpad sont analysées, y compris celles afférentes aux investissements immobiliers. Dans ce cadre se pose la question de l'impact d'investissements sur le prix de la journée. Aussi, pour éviter une augmentation trop importante du prix de la journée à la charge des résidents et de leurs familles, il est d'usage de lisser cette augmentation en anticipant, dès que la réflexion sur le projet est finalisée. Or la nomenclature comptable actuellement applicable aux Ehpad rattachés aux établissements publics de santé n'offre pas la possibilité de provisionner l'impact de ces évolutions tarifaires, se passe pour les établissements soumis à la nomenclature M22. Aussi, afin de sécuriser les investissements prioritaires pour la santé des résidents, une modification de l'instruction comptable est nécessaire. En effet, les départements, en leur qualité d'autorité de tarification, doivent pouvoir autoriser la constitution de provisions pour immobilisations et affecter un excédent réel d'exploitation à un compte spécifique qui pourra être repris lors de la réalisation des investissements. Dans mon département de la Drôme, six établissements sont concernés, dont, par exemple, l'Ehpad de Beauvallon géré par le centre hospitalier de Valence. Ce dernier, dont le plan

les Ehpad sont financés par l'assurance maladie au titre des prestations de soins, par le département au titre des prestations afférentes à la dépendance et par l'usager au titre de l'hébergement ou, à ce dernier titre, par le département lorsque le résident bénéficie de l'aide sociale Pour accueillir ces bénéficiaires, les Ehpad sont alors habilités par le département et le tarif afférent à l'hébergement est fixé par le président du conseil départemental. Il est déterminé en fonction des charges prévisionnelles de l'établissement.

sont prises en compte ; elles peuvent conduire à augmenter, à due concurrence, le prix de journée lié à l'hébergement. Afin de limiter la hausse des tarifs d'hébergement et le reste à charge que les investissements induisent pour les résidents, les arrêtés de 2008 et de 2014 relatifs aux instructions budgétaires et comptables M22 et M21 prévoient que les autorités de tarification peuvent verser aux Ehpad une allocation anticipée destinée à compenser les charges d'amortissement et les frais financiers liés à des opérations de rénovation ces crédits font l'objet d'une provision réglementée pour renouvellement des immobilisations. Ce dispositif vaut pour l'ensemble des Ehpad publics, que ces établissements relèvent du cadre budgétaire et comptable M21 ou M22. À cet effet, les instructions M21 et M22 prévoient un compte de « provision réglementée pour renouvellement des immobilisations Enfin, les Ehpad ont également la possibilité, dans le respect des dispositions prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé avec les autorités de tarification compétentes, d'affecter un résultat d'exploitation excédentaire en réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. Cette réserve est ensuite reprise pour compenser les charges d'amortissement induites par les nouveaux équipements de mise aux normes de sécurité. De même, cette réserve de compensation peut être constituée par l'ensemble des Ehpad publics, qu'ils relèvent des instructions M21 ou M22. Aussi les instructions M21 et M22 offrent-elles les mêmes possibilités aux Ehpad en matière de provisionnement et de financement des charges liées à des investissements. Cette analyse est partagée par la direction générale de la cohésion sociale.

de l'économie et des finances. Madame la secrétaire d'État, je souhaite appeler votre attention sur les dysfonctionnements des services postaux dans le département de l'Essonne. La situation devient de plus en plus inacceptable. En effet, depuis plusieurs mois, de nombreuses communes sont touchées par des difficultés liées à l'acheminement du courrier. Celles-ci sont régulières et l'exaspération de la population ne fait que s'accroître. C'est le cas d'Igny, de Bures-sur-Yvette, des Ulis, de Vert-le-Petit, du Coudray-Montceaux, de Bouray-sur-Juine, de Saintry-sur-Seine, de Saint-Chéron, entre Ces difficultés sont notamment des difficultés de gestion des ressources humaines, en particulier lorsque le personnel n'est pas remplacé pendant les vacances. À ces perturbations s'ajoutent les différents projets de modification des horaires d'ouverture de quelques bureaux et ceux, encore plus dommageables, de fermeture définitive, au sujet desquels les élus locaux demeurent, heureusement, pleinement mobilisés. Par Par ailleurs, il convient de préciser que ces situations ne sont pas sans conséquence pour les collectivités territoriales et pour les particuliers, sans oublier les acteurs économiques. À titre d'exemple, un chef d'entreprise se plaignait dernièrement de l'arrivée tardive de chèques qu'il attendait. Un administré m'a même écrit, la semaine dernière, pour me faire part des soucis qu'il rencontrait : à cause de l'arrivée tardive d'un courrier important, il a dû, à la dernière minute, commander un taxi, ce qui lui a coûté très cher, pour emmener son épouse dans un établissement de santé où elle avait été acceptée. En outre, l'envoi de lettres officielles et le soutien de parlementaires ne suffisant pas, des maires ont décidé d'agir en justice. Cette situation ne peut plus durer dans nos territoires. Le principe d'égalité, reconnu dans la Constitution, ne saurait être apprécié à géométrie variable. Plus que jamais, il appartient aux acteurs privés et publics de se mobiliser en faveur d'un service de proximité et de qualité, et ce sur l'ensemble du département. C'est pourquoi, devant l'ampleur de ce phénomène, je souhaiterais connaître les démarches que le Gouvernement engager, avec le groupe La Poste, pour mettre fin à cette situation et pour instaurer enfin une égalité de traitement entre les communes. La parole

En outre, le nombre de tournées à découvert s'est réduit. Selon La Poste, 32 des 35 sites de distribution du courrier du département de l'Essonne sont au niveau de qualité de service attendu. Trois sites, Palaiseau-Igny, Draveil et Brunoy, rencontrent encore des difficultés- il faut continuer à les accompagner - et font l'objet d'un soutien et d'un contrôle particuliers, afin de consolider les progrès constatés et de conforter le retour à la qualité du service et de la distribution. Plusieurs actions sont ainsi mises en oeuvre : le maintien des renforts en intérim pendant le temps nécessaire ; le déploiement progressif d'équipes de facteurs qualifiés pour réduire l'intérim et sécuriser la distribution ; le contrôle de l'efficacité des nouvelles organisations ; l'anticipation en 2019 des recrutements qui étaient prévus pour 2020, afin de porter à 9 les recrutements supplémentaires. S'agissant de la présence de La Poste dans l'Essonne, en 2018, l'offre de services postaux a globalement été renforcée et les horaires d'ouverture En outre, aucun bureau de poste situé en quartier prioritaire de la politique de la ville n'a été fermé, ces bureaux rendant des services essentiels aux habitants, notamment en matière d'accès aux services financiers de La Banque Postale. Mais vous avez raison, madame la sénatrice : ces difficultés sont inadmissibles et il faut y mettre un terme.

là ! La parole est à Mme Sylviane Noël, auteur de la question n° 960, transmise à M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. et du logement. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vivre et travailler en Haute-Savoie coûte cher, c'est une réalité qui pose aujourd'hui de sérieux problèmes pour le marché de l'emploi de ce département, tous secteurs d'activité confondus, publics comme privés. Avec plus de 10 000 nouveaux habitants chaque année en Haute-Savoie, il devient compliqué de maintenir certains services à la population, pourtant vitaux, par manque de candidats. candidats. Les agents qui arrivent du reste de la France renoncent au bout de quelques mois à rester en poste du fait du coût élevé de la vie, bien supérieur à la moyenne nationale. C'est principalement ce motif du « coût de la vie », notamment du logement, qui empêche les fonctionnaires et les salariés de s'installer durablement. Dans tous les secteurs d'activité, le taux de vacance de postes est critique, particulièrement dans la fonction publique hospitalière. La proximité avec la Suisse, notamment dans le Genevois et le Chablais, amplifie encore ce phénomène, en particulier pour les professions du secteur de la santé en raison de l'attractivité des salaires suisses. À l'heure où je vous parle, 181 lits d'Ehpad sont gelés dans le département, faute de personnel. L'octroi d'une prime de vie chère ou d'une indemnité de résidence en Haute-Savoie se révèle ainsi indispensable pour répondre au moins en partie à cette problématique. De même, il conviendrait de faire évoluer le zonage ABC affecté à de nombreuses communes de notre département, qui se révèle inadapté. Ce zonage prend en considération la tension du marché immobilier local comme critère de classement.

Bloquée en zone B2, la commune est ainsi privée de nombreuses aides à l'investissement locatif intermédiaire, notamment du dispositif fiscal de TVA à taux réduit qui s'applique aux logements intermédiaires portés par les investisseurs institutionnels en zone A et B1. Son caractère doublement frontalier, hautement touristique et très attractif d'un point de vue démographique fait incontestablement de la Haute-Savoie un territoire atypique. La mise en oeuvre d'un zonage et de dispositifs adaptés aux particularités de ce territoire est incontournable, et constitue un enjeu majeur pour le maintien des populations, le dynamisme économique et la vitalité des services publics. Je souhaiterais donc connaître les intentions du Gouvernement sur ces sujets. La parole

les communes qui mettent en place les opérations de revitalisation du territoire qui seront directement éligibles à ce dispositif. La réalité territoriale est avant tout connue par les élus locaux ou les agents qui travaillent

Je vous remercie,